Monsieur le Premier ministre, madame la vice présidente de l’Assemblée nationale,

Parlementaires, représentants de mouvements de la Résistance, de syndicats, de l’outre mer, puis de prisonniers et de déportés, tous incarnaient une parcelle de la légitimité française. Cette assemblée croyait de nouveau en l’avenir, après les heures les plus sombres, et alors que les combats continuaient dans certaines parties de notre territoire, en Alsace et autour des poches de l’Atlantique. Dans une France ruinée et meurtrie, l’espérance était plus que jamais présente au sein de cet hémicycle.

Marcel François Astier, Georges Bruguier, Pierre de Chambrun, Auguste Champetier de Ribes, Pierre Chaumié, Paul Fleurot, Justin Godart, Louis Gros, François Labrousse, Jean Odin, Joseph Paul Boncour, Marcel Plaisant, Camille Rolland, Henry Sénès. Et comment ne pas avoir aujourd’hui une pensée pour les sénateurs qui s’opposèrent à Vichy et au nazisme et qui furent assassinés, tels Marx Dormoy et Joseph Paul Rambaud. Dès le 25 octobre 1940, le général de Gaulle avait pris l’engagement solennel de rendre compte de ses actes aux représentants du peuple français, dès que celui ci aurait pu les désigner. Le 24 septembre 1941, cette assemblée provisoire prenait corps grâce à René Cassin, une ordonnance promulguée à Londres, qui disposait qu’il serait constitué une assemblée consultative destinée à fournir au Comité français de libération nationale (CFLN) une expression aussi large que possible de l’opinion française. Le 17 septembre 1943 est créée, à Alger, une Assemblée consultative provisoire chargée de préparer les institutions de la France après la Libération. Celle ci est uniquement consultative, ce qui ne l’empêche en rien de traiter de sujets essentiels, tels que l’effort de guerre, l’organisation future des pouvoirs publics en France, le vote des femmes.

femmes siégeront dans cet hémicycle en novembre 1944, auxquelles se joindront quatre femmes déléguées, à partir du 20 juillet 1945, au titre des prisonniers et déportés. Je tiens Lucie Aubrac, Madeleine Braun, Marie Couette, Claire Davinroy, Andrée Defferre, Alice Delaunay, Marthe Desrumaux, Annie Hervé, Marie Hélène Lefaucheux, Mathilde Péri, Gilberte Pierre Brossolette, Pauline Ramart, Marthe Simard, Marie Claude Vaillant Couturier, Marianne Verger et Andrée Viénot. Je revois

L’ordonnance signée le 21 avril 1944 par le général de Gaulle élargit le droit de vote aux femmes. Un an plus tard, le 29 avril 1945, alors que siège cette assemblée, les femmes ont pu voter pour la première fois lors des élections municipales. Le 12 juin 1945, l’Assemblée consultative provisoire adopte à l’unanimité une résolution permettant aux femmes d’exercer la fonction de magistrat. Le général de Gaulle dit lui même qu’« il serait vain […] de vouloir chercher un précédent historique à la création » de cette assemblée. Elle ne devait être qu’une étape vers le retour à des institutions démocratiques. L’Assemblée consultative provisoire délibère, mais ne légifère pas, puisqu’elle n’est pas issue du suffrage universel. Le général de Gaulle réserve au pouvoir exécutif, qu’il entend incarner, la faculté de procéder par ordonnances, lesquelles font l’objet de l’avis de cette assemblée. Une fois Paris libéré, il revint au secrétaire général de cette assemblée, Émile Katz Blamont, de chercher un lieu pour l’y accueillir : le Palais du Luxembourg fut choisi et remis en état en l’espace d’une semaine. Dès les jours qui suivirent le 25 août 1944, les fonctionnaires du Sénat, alors transférés rue Guynemer et boulevard Saint Michel, réintégrèrent le palais. consultative provisoire se réunit pour la première fois le 7 novembre 1944 sous la présidence de Paul Cuttoli, sénateur de Constantine. de Constantine. Dans du lendemain, on put lire : « Le Palais du Sénat a abrité la première séance de l’Assemblée consultative provisoire. C’était une minute émouvante que celle où nous avons revu, après des années de mort, cette salle illustre retrouver sa vie. » Au travers de cette assemblée, Charles de Gaulle veut retrouver tous les instruments de la légitimité démocratique et républicaine. Elle joua son rôle de représentation nationale, assura la continuité de la République et apporta au Gouvernement provisoire sa légitimité.

Attachée à l’unité de la Nation, après les divisions dévastatrices de la guerre, tout en étant respectueuse de la diversité, essence même de la démocratie, cette assemblée fut un lieu d’imagination, d’innovation, d’audace, de dialogue, d’écoute et de respect, dont l’exemple mérite d’être médité. Cette culture de la négociation et du compromis était déjà à l’ordre du jour dans une assemblée ne disposant pas de majorité préétablie, indispensable afin que le Gouvernement provisoire tienne compte de ses avis sur les sujets dont elle était saisie et des questions qu’elle soulevait dans le cadre des pouvoirs de contrôle dont elle disposait.

si cette union se crée, si elle se fortifie, alors nous aurons créé les conditions indispensables à une démocratie rénovée. » » Après une longue ovation, le général de Gaulle, alors président du Gouvernement provisoire, rendit hommage aux combattants de la première heure et aux Français qui les ont progressivement ralliés. Il rappela que, grâce à la Résistance, l’Assemblée consultative provisoire pouvait siéger au Palais du Luxembourg, symbolisant ainsi la continuité de la légalité républicaine dans une France encore en guerre. Pour le général de Gaulle, la réunion de l’assemblée consultative marquait « une nouvelle étape sur la route qui mène à la fois vers la victoire et vers la démocratie ».

De nombreux débats essentiels se déroulèrent en effet dans cet hémicycle. Dès le lendemain de l’intervention du général de Gaulle, un débat eut lieu sur la réintégration de l’Alsace Lorraine. Puis, dans les jours qui suivirent, se tint un débat sur la politique extérieure de la France, sur la question du ravitaillement, sur la reconstruction des réseaux de transport, sur l’organisation des armées. Ces débats furent aussi annonciateurs du processus de décolonisation et conduisirent cette assemblée à aborder l’avenir de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de l’Indochine.

obligeait la France à accompagner les aspirations de ceux qui, à leur tour, s’apprêtaient à prendre leur destin en main. Gaston Monnerville devint le président de la commission de la France d’outre mer de l’Assemblée

en février 1945 que l’assemblée consultative se consacra à l’examen des projets de budget des différents ministères, qui se poursuivit jusqu’au 31 mars. La déclaration de politique générale de Charles de Gaulle aura lieu le 2 mars, au milieu des débats budgétaires. Le général de Gaulle décida alors de venir présenter ses propositions de réforme des structures de l’économie nationale, et notamment les processus de nationalisation.

l’enrichira en abaissant le seuil des entreprises concernées à cinquante salariés. De même, lors de la séance du 31 juillet 1945, sera discutée la proposition de résolution de Gaston Tessier de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) sur l’organisation de la sécurité sociale. Le projet d’ordonnance visait à mettre en place l’organisation administrative amenée à assumer le service des différentes prestations. Je parlais d’une assemblée de la liberté retrouvée. Comment ne pas évoquer la séance exceptionnelle

Se tournant vers l’avenir, [la France] discerne le long et dur effort qui seul peut la rendre assez forte, fraternelle et nombreuse pour assurer son destin et, par là même, lui permettre de jouer pour le bien de l’Humanité un rôle dont il est trop clair que l’Univers ne se passerait pas.

fut celle de la liberté retrouvée. Comment ne pas évoquer également l’ordonnance du 18 novembre 1944 qui institua la Haute Cour de justice ? Lorsque s’ouvrit le 23 juillet 1945 le procès du maréchal Pétain, dix membres

cantonales, des élections à l’Assemblée constituante à la proportionnelle par département, et à la préparation d’une nouvelle Constitution. Le projet de Constitution française du 19 avril 1946, rédigé par la première assemblée constituante, prévoyait d’établir un régime parlementaire monocaméral, avec une assemblée unique élue au suffrage universel direct pour cinq ans. Ce projet fut voté par les députés le 19 avril 1946, mais les Français le rejetèrent lors du référendum du 5 mai 1946. Une nouvelle assemblée constituante fut élue le 2 juin. Celle ci rédigea un nouveau projet instituant un régime bicaméral, soumis lui aussi au référendum, qui fut adopté : il s’agissait de la Constitution du 27 Le Conseil de la République, né de cette Constitution, verra ses pouvoirs d’abord réduits par rapport à ceux du Sénat de la III République, mais il retrouvera ensuite la plupart d’entre eux.

Cette assemblée fut vraisemblablement un laboratoire pour la pensée du général de Gaulle. Elle fut pour lui un formidable poste d’observation de la vie politique française. Cette assemblée l’a ému,

et sous lequel [s’estompaient] trop souvent les intérêts supérieurs du pays ». Le général de Gaulle, lorsqu’il est revenu au pouvoir, a tiré la conclusion que la combinaison d’un exécutif puissant, responsable devant le Parlement, était une bonne formule de gouvernement.

notamment en faisant valoir, dans la confection des lois, les points de vue financier, administratif et local qu’une Assemblée purement politique [avait] fatalement tendance à négliger Au sein de cette assemblée, le général de Gaulle forgea ses convictions qui n’étaient « ni de gauche ni de droite » et qui n’avaient « qu’un seul objet qui est d’être utile au pays ». Mesdames, messieurs,

plus sûr, qui s’y exprima dans le mélange rare et exemplaire d’un devoir d’écoute, d’un respect mutuel et d’une volonté de recherche du consensus qui n’excluait en rien la fidélité aux convictions des uns et des autres. C’est, me semble t il, il, ce que le Parlement doit s’efforcer de faire aujourd’hui. Le bicamérisme est indispensable à l’équilibre de nos institutions, particulièrement dans le moment politique que nous vivons.

Il est […] facile de comprendre pourquoi il faut à la France une puissante deuxième chambre […]. Notre régime électoral nous empêche de connaître les majorités cohérentes qui assurent, sans règles détaillées, la bonne marche du régime parlementaire. prescience que nous vivons concrètement. Oui, je suis convaincu que le bicamérisme est utile pour notre démocratie. Le Sénat d’aujourd’hui,

oser expérimenter, oser être audacieux, oser en même temps assurer la stabilité de l’essentiel. Le Sénat souhaite réconcilier la France avec ses territoires en donnant plus de liberté, de stabilité, de confiance et de respect aux élus.

Ce moment solennel nous invite à honorer l’héritage de ceux qui, voilà quatre vingts ans, se sont installés ici, au Palais du Luxembourg, dans un contexte de guerre, au cœur d’un pays profondément meurtri, fracturé, divisé. Le 7 novembre 1944 s’ouvrait la première séance de l’Assemblée consultative provisoire. Ce fut l’un de ces instants fondateurs jalonnant notre histoire parlementaire et un acte symbolique puissant, marquant la renaissance démocratique de la France. Au travers de cette assemblée, notre nation, par le courage et la détermination de ses représentants, commença à se reconstruire dans la légitimité républicaine. Ces femmes et ces hommes venus de la Résistance, du monde syndical, de la société civile portaient la voix de la liberté et le refus de la tyrannie. Ils sont pour nous un exemple éternel de résilience et d’engagement républicain. Le choix d’installer l’Assemblée consultative provisoire au Palais du Luxembourg n’était pas anodin ; il constitua un acte de foi envers la démocratie parlementaire. Ce palais, notre Sénat, représentait depuis longtemps la continuité des institutions de la République. En y plaçant cette assemblée, le gouvernement provisoire du général de Gaulle signifiait à la Nation que la République n’avait jamais cessé d’exister, même sous la pression des forces d’occupation et du régime de Vichy. Dans ces murs, la démocratie renaissait de ses cendres, portée par la foi en des valeurs auxquelles nous croyons plus que jamais : l’unité, la souveraineté et le respect des institutions. Cette assemblée était, à l’image de la nôtre, synonyme de diversité. Elle réunissait des parlementaires en exil, des représentants de mouvements de la Résistance, des syndicalistes, des personnalités de tous horizons politiques et sociaux. Ensemble, ils ont incarné une France unie, par delà les désaccords partisans. À l’heure où notre pays fait face à plusieurs défis de taille, nous devons plus que jamais avoir en tête que les différences idéologiques n’empêchent pas les compromis. Cette capacité à trouver un terrain d’entente au service de l’intérêt général doit, je le crois, plus que jamais demeurer au cœur de l’action du Sénat. Au delà du symbole et des idéaux qu’elle a portés, l’Assemblée consultative provisoire a marqué une nouvelle étape sur la route qui mène à la fois vers la victoire et vers la démocratie. Elle a porté des réformes profondes en matière sociale et économique, en lien avec les aspirations du Conseil national de la Résistance. Elle a soutenu les bases d’une protection sociale solide, le droit au travail et à la sécurité, l’accès à la santé et à l’éducation pour tous. Elle a travaillé à rendre la France plus juste et plus solidaire et à inscrire dans la loi les droits et les protections pour lesquels ses membres s’étaient tant battus. Ces réformes constituent le fondement de notre modèle social et doivent être préservées. Par ses travaux, l’Assemblée consultative provisoire porta également un message de souveraineté et d’indépendance. La France de 1944 voulait réaffirmer sa place sur la scène internationale, retrouver son honneur et montrer au monde que, même affaiblie,

Nous devons continuer de défendre une France maîtresse de ses choix, forte de ses institutions et fidèle à ses valeurs républicaines. L’histoire de cette assemblée nous rappelle enfin que la responsabilité de gouverner est indissociable de celle de représenter le peuple. de leurs travaux, les membres de l’Assemblée consultative provisoire ont démontré une humilité exemplaire, une écoute, un sens du devoir que nous devons continuer de faire vivre. Ils ont rappelé que la légitimité politique trouve sa source dans l’engagement pour le bien commun et dans le respect de nos concitoyens. À l’heure où la défiance à l’égard de nos institutions grandit, où le lien de confiance entre les citoyens entre les citoyens et leurs représentants s’érode, nous avons le devoir de renouer avec cette exigence démocratique. Comme le disait André Malraux, la France n’est grande que lorsqu’elle se bat pour les idéaux de la République. C’est ce combat qui doit inspirer qui doit inspirer notre travail et notre engagement. Mes chers collègues, en célébrant cet anniversaire, nous honorons un prestigieux héritage. Par cet acte, nous rendons hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont cru en la France, dans l’honneur et l’indépendance. Souvenons nous que nous portons, dans cet hémicycle, une responsabilité immense : celle de faire vivre cet héritage et de le transmettre. C’est là notre devoir envers le peuple français. La parole

j’ai très mal tourné. Par cette cérémonie, nous célébrons avec force les lueurs d’espoir qui ont été ravivées après les heures les plus sombres de notre histoire. Après le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944, au moment de la libération progressive de la France, la question de la gouvernance du pays après la chute du régime de Vichy est devenue cruciale. Le Gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle, a alors été créé pour organiser la transition entre l’occupation allemande et le rétablissement de la République. L’Assemblée consultative provisoire a été conçue dans ce contexte si sensible, si particulier pour l’histoire de la France. Elle était opportunément

place. Sa principale attribution était de formuler des avis sur les questions les plus délicates que le gouvernement français avait à trancher autour de la reconstruction économique et politique du pays après les ravages causés par la guerre.

les 80 ans de l’installation de cette assemblée dans nos murs revêt une dimension particulière dans le contexte politique mondial si instable, pour ne pas dire dangereux, que nous connaissons.

général de Gaulle lors de la première réunion de cette assemblée, le 9 novembre 1944. C’est donc ici qu’il choisit de célébrer la victoire au lendemain de la capitulation allemande de mai 1945.

la souveraineté du peuple ». Sûrement du fait de la méfiance envers le parlementarisme d’avant guerre, cette assemblée n’avait pas non plus de vocation législative : vous le savez, elle n’était que consultative. D’ailleurs, les historiens ont rappelé que le président du gouvernement provisoire était libre de tenir compte ou non des avis émis ; manifestement, il ne s’en est pas privé.

Les discussions qui ont animé l’Assemblée consultative provisoire ont préparé de grandes réformes : la création de la sécurité sociale ; l’instauration d’une véritable démocratie sociale contribuant à l’amélioration des conditions de vie matérielles et à la dignité des travailleurs ; la libération de la presse ; la définition d’une nouvelle politique de la jeunesse ; ou encore la proposition d’accorder le droit de vote aux femmes, dès les premières élections d’après guerre. À ce propos, je tiens à préciser que douze femmes

chers collègues, le Palais du Luxembourg a donc été l’écrin de la liberté retrouvée, pour reprendre l’une des expressions de notre président.

le 7 novembre 1944, lorsque l’Assemblée consultative provisoire se réunit pour la première fois à Paris, le drapeau nazi flotte encore sur Strasbourg. À cette date, Metz, les Vosges, l’Alsace et la Lorraine sont encore sous contrôle allemand. Le 7 novembre 1944, la guerre n’est donc pas finie, loin de là, mais les forces de la Résistance tiennent à placer le plus tôt possible la France libérée sous le signe de la démocratie. Tel est le sens de l’installation de cette instance ici même, au Palais du Luxembourg.

ni une invasion étrangère ni une dictature collaborationniste n’ont pu venir à bout de notre attachement à la démocratie. Deuxièmement, l’Assemblée consultative provisoire est une assemblée représentative. En l’instaurant, le général de Gaulle réaffirme l’engagement de la France à bâtir la démocratie sur le socle de la représentation nationale. Troisièmement, permettez moi de le dire dans un clin d’œil avec une pointe de facétie, en nous réunissant aujourd’hui, nous célébrons aussi le fait que, désormais, les assemblées ne soient plus ni provisoires ni consultatives…

Dans l’esprit du Général, cette dernière est « un exutoire » au « bouillonnement » des forces politiques disparates qui ont contribué à la victoire de la France – toute ressemblance avec la situation actuelle est évidemment fortuite… Pour autant, cette assemblée joua un rôle non négligeable dans la reconstruction républicaine : réintégration de l’Alsace Lorraine, construction européenne, reconnaissance de l’éphémère alliance franco soviétique, réorganisation des transports, désignation des des juges de la Haute Cour de justice, nationalisations, réforme fiscale… Les dossiers les plus brûlants du moment lui furent soumis. En tant que président du groupe Union Centriste, vous me permettrez d’évoquer brièvement quelques figures marquantes de cette époque, en commençant par Maurice Schumann. Cofondateur du Mouvement républicain populaire (MRP), celui ci s’est illustré par sa vision d’une Europe fondée sur la coopération et une paix durable. Il a porté haut cet idéal au sein de la commission des affaires étrangères, et son message résonne encore à l’aune des défis européens

Marie Hélène Lefaucheux, résistante et pionnière, qui s’est illustrée dans l’aide au rapatriement des déportés. Parmi les premières femmes à devenir parlementaires, elle s’est battue avec ardeur pour les droits des femmes. Au sein de la Commission de l’équipement national, de la production et des communications, parmi les représentants de l’Organisation civile et militaire (OCM) et, plus tard, à l’ONU, où elle a présidé pendant dix ans la Commission de la condition de la femme, elle a défendu l’idée d’une juste place des femmes dans la vie publique. Nous devons faire perdurer sa volonté en promouvant une politique d’intégration plus paritaire. Enfin, je rendrai hommage à André Colin, qui fut le premier président de notre groupe, de 1963 à 1971. Homme de dialogue, il a joué un rôle au sein des commissions de la jeunesse et des sports, de l’intérieur et de la santé publique et du règlement de l’Assemblée consultative provisoire, proposant des mesures pour les aides aux familles, le remembrement agricole et le développement des régions – des engagements qui restent un modèle pour nous aujourd’hui. Je le disais en préambule, le fait de commémorer est l’occasion d’honorer la mémoire, mais aussi de mesurer le chemin parcouru pour éclairer les temps présents. Le défi du 7 novembre 1944 était le retour du parlementarisme ; quatre vingts ans après, le défi du 7 novembre 2024 est peut être de le réinventer. consultative provisoire, l’Assemblée constituante a élaboré la Constitution de la IV République, qui périt en 1958 de son incapacité à assurer une stabilité institutionnelle suffisante. Et voici qu’aujourd’hui la Constitution de la V République, référence s’il en est du parlementarisme rationalisé, confronte de nouveau notre pays à une majorité au socle commun fragile. Il est loin le temps où certains voulaient faire disparaître le Sénat. de le souligner le président Larcher, le bicamérisme a démontré sa raison d’être. Pour que nos assemblées ne soient pas de nouveau réduites au rang d’exutoire au bouillonnement des forces politiques, il nous appartient individuellement de répondre, en responsabilité, aux attentes que la situation nous impose. Mais il est aussi de notre responsabilité collective de réfléchir aux adaptations nécessaires,

tenait sa première séance de travail au Palais du Luxembourg. Je n’en ai certes aucun souvenir, mais je me rappelle la reconstruction de notre pays ; c’est mon enfance. Je me souviens que la France entamait alors, dans la douleur, la décolonisation. Il y avait encore des bidonvilles dans notre pays. Je me souviens que l’Europe, autrefois si orgueilleuse, découvrait, au petit matin, la honte : celle des ravages de la Seconde Guerre mondiale, des crimes atroces, des camps de concentration, des exécutions sommaires, de la Shoah, des brigades de la mort, de la collaboration des autorités locales et, en ce qui nous concerne, nationales. Et pourtant, il soufflait un vent d’optimisme et d’enthousiasme sur le pays. La reconstruction est une période dont on parle peu en France, marquée par les stigmates de la IV République et par le réveil paradoxal de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : à la fois dans le camp des vainqueurs et humiliée par la défaite militaire et morale que notre pays a connue en 1940. Pourtant, la reconstruction est aussi la période où la France, en repartant de très bas, a réussi à redevenir une puissance mondiale respectée. Malgré l’instabilité ministérielle et le début de la guerre froide, l’Assemblée consultative provisoire a su poser les bases d’un pays fort d’une construction européenne visant à bannir la guerre de notre continent et à construire une prospérité commune. Devant les difficultés d’approvisionnement qui frappaient les Français au quotidien, le Gouvernement a réussi à relancer rapidement et efficacement la production et les chaînes logistiques. Face à l’inflation galopante, Antoine Pinay a su assainir en seulement dix mois les finances publiques et stabiliser le franc, engendrant une hausse massive du pouvoir d’achat des Français. J’ai connu cette époque, et je peux témoigner que les débats politiques étaient au moins aussi enflammés qu’actuellement, si

forte qu’auparavant. Au cœur des crises, l’esprit français ne se penche pas uniquement sur le meilleur moyen d’abattre son ennemi, il est résolument tourné vers l’avenir. C’est dans la Résistance, par l’union de la rose et du réséda, qu’est née l’Assemblée consultative. Dans ce pays

C’est dans les caves, dans les greniers, à l’abri des miliciens et des soldats allemands que l’armée des ombres imaginait l’organisation des pouvoirs, de la santé, de la vie économique de notre pays après la victoire. Ainsi, le 15 mars 1944, huit mois avant la séance inaugurale de l’Assemblée consultative que nous commémorons aujourd’hui, le Conseil national de la Résistance signait son programme d’action. Alors que le débarquement de Normandie n’avait pas encore eu lieu, alors qu’ils préparaient les échéances militaires à venir, ses membres avaient à cœur de dire comment il fallait rétablir nos institutions et notre démocratie, comment devrait fonctionner la vie dans les entreprises et dans la société.

les crises qui se profilent à l’horizon menacent sérieusement notre pays dans toutes ses dimensions : notre économie, notre cohésion sociale, l’environnement dans lequel nous vivons. Et je n’oublie pas que la guerre fait de nouveau rage sur notre continent… Cette cérémonie est l’occasion de rappeler qu’aussi grandes soient les difficultés,

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la vice présidente de l’Assemblée nationale, mesdames, monsieur le premier enjeu d’une commémoration est de tirer la leçon des événements que nous commémorons. C’est ce que faisait, le 9 novembre 1944, le général de Gaulle en résumant les années tragiques qui ont précédé la libération de la France

ans plus tard, il est à craindre que la France et, plus généralement, les démocraties n’aient oublié ces enseignements et l’aveuglement devant les totalitarismes que dénonçait de Gaulle.

incapables de convaincre leur peuple qu’il fallait les combattre tant qu’il était encore temps. Ils avaient une excuse : ils étaient confrontés pour la première fois à l’essor des régimes totalitaires, pire encore, à leur improbable alliance. Nous n’avons plus cette excuse. Sous nos yeux l’histoire du XX siècle se répète au XXI siècle. Aux totalitarismes nazi et soviétique ont succédé les dictatures russe, chinoise, nord coréenne et iranienne, et au pacte germano soviétique l’alliance de ces quatre tyrannies. À l’Anschluss, aux Sudètes et à la Pologne répondent l’invasion de la Géorgie et de l’Ukraine, les menaces sur la Moldavie, sur Taïwan et toute la mer de Chine et les appels à la destruction d’Israël. À l’obsession d’Hitler et de Staline de détruire par tous les moyens l’ordre démocratique fait suite la guerre que les despotes actuels ont ouvertement déclarée au monde de paix, de liberté et de prospérité instauré par les démocraties en 1945. Aux cinquièmes colonnes qu’étaient les partis communistes et fascistes de l’entre deux guerres en Europe ont succédé des populismes d’extrême droite et d’extrême gauche ouvertement alliés aux tyrans.

À force de détester leur pays, les extrémistes finissent toujours par le trahir. Beaucoup de nos dirigeants affirment que nous ne sommes pas en guerre contre l’internationale des dictateurs, comme Daladier rentrant de Munich se félicitait d’avoir sauvé la paix. paix. Il n’y a rien de plus dangereux que de croire que nous ne sommes pas en guerre contre des gens qui sont en guerre contre nous et qui le disent. L’Europe doit comprendre qu’il est urgent pour elle de redevenir une puissance militaire

les Français ont fait tout ce qui était nécessaire pour mener à la guerre, parce qu’ils en avaient peur », disait Raymond Aron. Il ajoutait : « Je crois à la victoire des démocraties, à condition qu’elles le veuillent.

Or les Occidentaux continuent d’interdire aux Ukrainiens d’utiliser leurs missiles pour frapper en Russie les bases d’où partent les avions et les bombes qui détruisent l’Ukraine. La dissuasion nucléaire est censée sanctuariser notre territoire et préserver notre liberté d’action c’est au nom de cette même dissuasion que nous théorisons notre inaction, que nous laissons à Poutine le monopole de la menace et de l’agression. Nous savons pourtant que ses alliés chinois lui interdisent son emploi. Son abstention après que les Ukrainiens ont franchi la frontière russe à Koursk apporte la preuve que ses lignes rouges ne sont qu’un bluff. La Seconde Guerre mondiale, disait de Gaulle le 9 novembre 1944, a eu pour cause « la frénésie dominatrice d’un système politique, social, moral, abominable […], mais revêtu du sombre attrait de la puissance. Elle a trouvé, pour la favoriser, la dispersion des États du parti de la liberté […], les divisions passionnées, les routines de tous ordres, la défaillance des élites dirigeantes En cet anniversaire, alors que les Ukrainiens meurent chaque jour par milliers pour défendre notre liberté, dans une indifférence chaque jour croissante, chaque jour plus préoccupante, puissions nous méditer ces paroles prophétiques. La parole

C’est le général de Gaulle lui même qui, le 9 novembre 1944, inaugura les travaux de cette assemblée dont la constitution marquait la renaissance de la démocratie. Il faut se transporter dans le temps, en cet automne de 1944 ; imaginer la situation de notre pays, de l’Europe et même du monde entier, confronté à une violence inouïe.

Emmanuel d’Astier de La Vigerie, Maurice Schumann, Daniel Mayer, Lucie Aubrac, Robert Chambeiron, Pierre Cot et tant d’autres, siégeaient communistes : André Mercier, membre du Conseil national de la Résistance, Georges Cogniot, Jacques Duclos, Léo Figuères, Benoît Frachon ou encore Waldeck Rochet. L’Assemblée consultative provisoire s’est fixé pour objectif la sortie des années noires, le redressement du pays et la marche vers les jours heureux, auxquels aspire

C’est le programme du Conseil national de la Résistance qui est au cœur des débats de cette assemblée et de ses décisions. Ce programme – il faut le rappeler – porte en germe le retour de la démocratie et de la justice sociale.

ceux qui ont sauvé la démocratie, qui ont porté l’idée de justice au plus haut. Mon regard s’est arrêté sur le nom de Mathilde Péri, épouse de Gabriel Péri, journaliste

la Résistance, ô combien exemplaire, incarnée par Jean Moulin et tant d’autres hommes et femmes héroïques ; celles des débarquements alliés, à la fois extraordinaires et essentiels à la libération de la France. Bien sûr, le visage de l’espoir, c’est aussi celui du général de Gaulle, refusant farouchement la défaite et déclarant depuis Londres le 18 juin 1940 : « Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Par leur audace, ces quatre vingts parlementaires rendent un peu de fierté à leur pays défait. Le 10 juillet 1940, au sein du groupe de la Gauche démocratique, l’honneur est du côté des sénateurs Camille Rolland, Jean Odin et François Labrousse, parmi d’autres.

aussi de l’épopée de cette France en marche pour la liberté, comme le Gouvernement provisoire de la République française, qui succéda au Comité français de libération nationale. Bien que tournés vers la reconquête par les armes, les acteurs de la France libre n’ont pas oublié la nécessaire reconquête des institutions par le rétablissement, en 1943 à Alger, d’une assemblée parée autant que possible de la légalité républicaine.

le contexte politique de cette semaine donne à notre séance une tonalité plus solennelle encore. Hier tombait en effet le verdict dramatique de l’élection présidentielle américaine. le peuple souverain a choisi pour conduire les destinées de la Nation un homme qui, entre autres outrages, s’est rendu complice, si ce n’est coupable, d’une tentative de coup d’État contre un Parlement lui Le scrutin de mardi dernier est venu rappeler que les démocraties sont mortelles et que, souvent, elles se donnent elles mêmes la mort. À l’heure où nous craignons l’effondrement de l’une des plus grandes et plus vieilles démocraties du monde, d’une démocratie qui en a inspiré tant d’autres à travers l’Histoire,

Je ne crois pas que le Gouvernement provisoire de la République française et l’Assemblée consultative provisoire se soient contentés de rétablir la légalité républicaine. Je crois qu’ils ont pavé le chemin du rétablissement de la République tout entière. Les héritiers du gaullisme et les constitutionnalistes débattront encore longtemps de cette question. Mais je suis de ceux pour qui la III République est morte le 10 juillet 1940

Par conviction personnelle sans doute, par nécessité politique certainement, le général de Gaulle n’a pas souhaité proclamer la République au balcon de l’Hôtel de Ville, comme l’avait fait Gambetta en son temps. la République n’avait jamais cessé d’être et il a tout fait, en pleine guerre, pour en rétablir les institutions. Dès l’instauration du Comité national français (CNF), premier gouvernement de la France libre, le 24 septembre 1941,

Je ne suis pas certain que le général de Gaulle ait été un grand défenseur du parlementarisme ; mais il était indubitablement un grand défenseur de la République, régime dont le principe constitutif est la séparation des pouvoirs, notamment législatif et exécutif.

C’est notamment cette construction institutionnelle originale, cette « surprenante aventure », pour reprendre les termes d’Émile Katz Blamont, secrétaire général de l’Assemblée consultative provisoire, qui a permis au Général de convaincre Roosevelt de ses intentions républicaines et à la France d’éviter l’occupation par les troupes alliées. Tel n’est toutefois pas le seul mérite de cette assemblée,

Durant deux ans, dans un esprit de concorde républicaine entre les représentants des partis et mouvements de Résistance de gauche et de droite, unis contre l’extrême droite de Vichy, l’Assemblée consultative provisoire a accompagné le Comité français de libération nationale, puis le Gouvernement provisoire de la République française, dans la mise en œuvre du programme du Conseil national de la Résistance : conduite des opérations militaires et de la politique de défense ; réorganisation des pouvoirs publics ; création création des comités d’entreprise ; et surtout préparation des grandes réalisations du GPRF après la victoire, parmi lesquelles la nationalisation de grandes banques et d’entreprises stratégiques, l’instauration de la sécurité sociale, l’encadrement des prix des denrées alimentaires et la préparation de la Constituante. Monsieur

pour reconstruire une République plus démocratique, conduire une politique économique résolument administrée, instaurer une politique sociale historiquement ambitieuse, que nous chérissons encore aujourd’hui, et accompagner judicieusement un vent de modernisation de la société.

de nombre d’anciens membres de la Haute Assemblée ainsi que de représentants des organisations syndicales et du président de la fondation Charles de Gaulle. Monsieur le président, j’ai été très touché de votre invitation.

du 7 novembre 1944 est d’abord un symbole démocratique. Paris a été libéré le 25 août. Strasbourg sera reprise le 23 novembre.

de la légalité et des institutions républicaines. Le Gouvernement provisoire de la République française s’est installé à Paris le 31 août 1944. L’Assemblée consultative provisoire vient quant à elle préfigurer le retour de la vie parlementaire.

lequel vient rendre compte des grandes étapes du rétablissement de la légalité républicaine. À la fin du mois de juillet 1945, cette assemblée, unique en son genre, avait rempli sa mission.

Il était alors temps de passer la main à une assemblée constituante. Pour paraphraser le général de Gaulle dans sa déclaration du 12 juillet 1945, la Nation pouvait « reprendre en main ses destinées